le 5 mars dernier, nous examinions ma proposition de loi qui faisait suite au drame de la rue d'Aubagne à Marseille, drame qui a marqué durablement les esprits, tant il a cruellement endeuillé huit familles puis entraîné l'évacuation de plusieurs milliers de personnes.

doit être à la mesure du drame pour que plus jamais nous n'ayons à revivre cela. Aujourd'hui, il nous faut faire plus, plus vite et plus efficacement. Lutter contre l'habitat indigne est notre affaire à tous : il s'agit d'une priorité nationale. Je suis très satisfait que le Sénat ait pu s'emparer de ce sujet, car, comme l'a constaté la commission des affaires économiques lors de ses déplacements, les élus, et les maires en particulier, sont très impliqués et engagés dans la lutte contre l'habitat insalubre. sont pourtant trop souvent freinés dans leurs actions, empêchés dans d'autres cas, du fait de la complexité des procédures, de la diversité des autorités concernées et de l'enchevêtrement des compétences en matière de logement indigne. Il nous revient de lever les freins constatés pour que la lutte contre l'habitat insalubre soit plus rapide et plus efficace. Je remercie la commission des affaires économiques du bon accueil fait aux propositions que j'ai exposées dans ce texte, examiné une première fois en mars dernier. Vous avez souhaité, madame le rapporteur, prendre davantage de temps pour approfondir la réflexion sur les dispositifs que nous avions proposés au travers des neuf articles visant à renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales, accélérer les réponses aux situations d'insalubrité et renforcer les sanctions à l'encontre des marchands de sommeil. Les nombreuses visites de terrain, ainsi que les auditions auxquelles vous avez procédé à Montfermeil, à Marseille, dans la Somme, en Guadeloupe, en Martinique, pour ne citer que ces déplacements, ont permis d'appréhender très concrètement des situations multiples qui appelaient des réponses ciselées, des dispositifs les plus ajustés possible, sans pour autant pénaliser un secteur.

Je compte, nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour nous épauler et compléter ce qui doit l'être, afin de faire avancer rapidement la lutte contre l'habitat insalubre, et notamment d'accompagner en moyens humains, financiers et d'ingénierie ce chantier législatif majeur. Les travaux de votre commission, madame la présidente, ont validé les principales orientations défendues par Mme le rapporteur à l'aune des observations collectées sur le terrain, celle-ci nous présentera dans quelques instants. L'une des dispositions que j'approuve pleinement est la mise en place d'une police spéciale du logement qui traitera, selon une procédure identique, l'ensemble des cas cas d'habitat dégradé, qu'il soit en péril, insalubre, indigne ou indécent. Il s'agit là d'une mesure de simplification de premier plan,

et les collectivités. Le traitement des logements en péril et celui des logements insalubres demeureront donc distincts pour le moment : le maire continuera de prendre des arrêtés de péril et le préfet continuera de prendre des arrêtés d'insalubrité.

ou d'insalubrité, tout en donnant un droit de priorité aux collectivités territoriales qui souhaiteraient profiter du bien exproprié. Vous accentuez les sanctions que nous proposions à l'encontre des marchands de sommeil en sorte que les collectivités territoriales bénéficient du produit des amendes prononcées par le préfet pour non-respect des règles relatives au permis de louer. louer. Madame le rapporteur, vous appelez tous les acteurs à se mobiliser pour lutter contre l'habitat indigne. Je ne peux que partager pleinement cette volonté. Il nous faut être à la fois inventifs et concrets dans les dispositifs que nous proposons, à l'image du parcours de rénovation énergétique performante de la ville de Montfermeil où je me suis rendu, moi aussi, en février dernier.

La deuxième ville de France doit pouvoir se doter d'un projet urbain global plus dynamique. Cette volonté ne peut se concrétiser sans le concours de ses habitants et de ses commerçants, que nous devons associer et faire revenir, Parvenir à lutter contre la spirale négative de la dégradation du bâti et, par suite, des conditions de vie suppose une approche transversale et coordonnée des actions à mener : plan de sauvegarde, projet urbain, suivi des relogements, accompagnement social et, bien sûr, lutte contre l'habitat indigne. Ainsi, et pour aller plus loin, on peut penser que la mise en oeuvre d'une opération de requalification des copropriétés dégradées serait susceptible d'apporter une aide massive aux petits propriétaires privés qui font face à la dévalorisation de leur immeuble et du quartier sans avoir les moyens financiers d'y remédier efficacement. Plus largement encore, il serait opportun de créer une zone franche urbaine dans le centre de Marseille, afin d'impulser une nouvelle dynamique économique et sociale. Celle-ci prendrait la forme d'un double panel d'aides et de subventions cumulatives, afin que ce périmètre puisse renouer avec l'attractivité et la réussite économique. Le retour de petites entreprises et du commerce de proximité contribuerait à la rénovation du centre-ville en engageant un processus de requalification des réseaux, de réhabilitation des devantures commerciales des façades d'immeubles, de rénovation des locaux professionnels, associé à l'utilisation des nouveaux outils destinés à lutter contre l'habitat indigne. Telles sont les prémices à l'instauration d'un cercle vertueux qui redonnera

aussi que l'Assemblée nationale se saisisse du texte sans tarder. C'est un combat commun que nous devons mener ensemble pour qu'il aboutisse rapidement, car c'est une vision de la dignité de l'homme que nous partageons assurément sur toutes les travées ! La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, il y a sept mois, plusieurs immeubles s'effondraient rue d'Aubagne à Marseille entraînant la mort de huit personnes et obligeant plus d'un millier d'habitants à quitter leur logement. Cet événement dramatique nous faisait prendre conscience, s'il en était besoin, de la situation de l'habitat indigne dans l'ensemble de nos territoires, urbains comme ruraux. La proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, déposée par notre collègue Bruno Gilles, nous a permis de revenir sur ce sujet- ô combien important ! -de l'habitat indigne. En mars dernier, nous avons décidé de prendre plus de temps pour approfondir l'examen de ce texte. Il s'agissait d'examiner d'autres dispositifs de prévention et de simplification des procédures en matière d'habitat indigne. Je remercie Bruno Gilles d'avoir compris le sens de notre démarche. Nous avons cherché les moyens de lever les freins législatifs à une mise en oeuvre efficace de cette politique. Le texte établi par la commission, que nous examinons ce soir, tient compte des observations recueillies lors de nos nombreux déplacements et auditions. Les principales orientations retenues par Bruno Gilles ont ainsi été confortées. La commission a centré ses propositions autour de quatre axes. La détection et la prévention de l'habitat indigne constituent un axe essentiel que l'on néglige bien trop souvent. Or c'est bien connu : « Mieux vaut prévenir que guérir. » Plus on intervient en amont, plus on limitera le nombre de logements indignes. La commission a ainsi créé un chapitre spécifique dans la proposition de loi qui comprend deux mesures. La première concerne le diagnostic technique global, qui permet de faire un état des lieux de la copropriété. L'outil est intéressant à un double titre. Les copropriétaires bénéficient d'un bilan qui leur sert de base pour engager des travaux. Il s'agit également d'une source de données pour les élus. À Aubervilliers, nous avons vu des immeubles dont la façade est impeccable, mais dont l'intérieur est, en réalité, dans un état de dégradation avancée.

La seconde mesure concerne les syndics professionnels. Ils sont aux premières loges pour détecter les logements indignes. La commission leur a donné la possibilité à des signalements dans les cas d'habitat insalubre, dangereux et indécent, sans que l'on puisse leur opposer le principe de confidentialité des données.

d'une police spéciale du logement. La multiplication des polices n'est pas un gage d'efficacité et peut aussi être source de contentieux. Les événements dramatiques de Marseille nous ont rappelé l'urgence d'agir. Monsieur le ministre, le délai de dix-huit mois dont dispose le Gouvernement pour réformer ces polices par ordonnances est bien trop long. Nous devons arrêter de tergiverser ! C'est pourquoi la commission a décidé de revenir sur l'habilitation à légiférer et de modifier directement le droit en vigueur.

ou le maire lorsque ce dernier souhaite conserver ses pouvoirs de police, l'État demeurant compétent en cas de carence. Enfin, cette police spéciale a vocation à suivre une procédure identique dans tous les cas. Malheureusement, Bruno Gilles l'a rappelé, l'article 40 de la Constitution empêche tout transfert de compétences et nous empêche donc de proposer cette réforme dans sa globalité. C'est bien dommage. Je ne peux à ce stade que demander au ministre d'engager cette réforme dans les délais les plus brefs. Le traitement des logements en péril et celui des logements insalubres demeurent donc distincts à ce stade. Le maire continuera de prendre des arrêtés de péril et le préfet continuera de prendre des arrêtés d'insalubrité. Mais, dans les deux cas, ils devront suivre une procédure qui, elle, sera identique. Bruno Gilles a proposé d'améliorer deux étapes de la procédure : la phase d'instruction et la phase de relogement. S'agissant de la phase d'instruction, la commission est allée dans son sens. Elle a donné un délai global de deux mois, à la fois pour visiter les locaux et transmettre le rapport à la personne concernée. Elle a également accéléré la phase de relogement en cas d'interdiction définitive d'habiter, tout en tenant compte du marché du logement. Aussi le délai maximal est-il fixé à six mois dans les zones tendues et à trois mois dans les zones non tendues. Le dispositif devra certainement être amélioré. Il s'agit de la première pierre de l'édifice. Au Gouvernement, là encore, de démontrer sa volonté d'agir et d'apporter des modifications complémentaires. Malgré leur volontarisme, les maires sont souvent désarmés, faute de disposer des outils adéquats. Bruno Gilles a proposé d'octroyer de nouveaux pouvoirs aux élus locaux pour mieux lutter contre l'habitat indigne. dite loi ALUR, et de la loi ÉLAN, nous avons cherché à améliorer le régime juridique des permis de louer et de diviser. Bruno Gilles proposait que le silence gardé pendant deux mois vaille rejet de la demande. Les professionnels sont partagés et les effets de cette mesure sont incertains.

Les communes peuvent être découragées face à l'ampleur de la tâche que représente l'instruction des permis de louer. La commission a décidé que le bailleur serait dispensé de cette procédure lorsqu'il a bénéficié, pour le bien concerné, d'un permis de louer depuis moins d'un an. devra cependant informer la collectivité de la mise en location du bien. De nombreux élus sont confrontés à des propriétaires qui n'exécutent pas les travaux définis

de soumettre à la procédure dérogatoire d'expropriation les immeubles qui font l'objet d'une interdiction définitive d'habiter et dont le propriétaire n'a pas réalisé les travaux. Elle a néanmoins ajouté des critères pour rendre le dispositif recevable au regard du droit de propriété. Les collectivités sont bien souvent à l'origine du signalement de l'insalubrité ou du péril. Elles sont mieux à même que l'État de valoriser et de gérer un bien exproprié sur leur territoire. Ça dépend ! Aussi la commission leur a-t-elle donné un droit de priorité pour bénéficier du bien en péril ou insalubre exproprié. De même, la commission a jugé intéressante l'idée de mettre en place un droit de préemption adapté à la lutte contre l'habitat indigne. Elle n'a pu pas le faire, là encore, là encore, en raison du pouvoir limité du Parlement en matière d'initiative financière. C'est cela le parlementarisme rationalisé que l'on voudrait pourtant encore renforcer a néanmoins proposé que le nom de l'acquéreur soit mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, ce qui permettra aux collectivités d'avoir accès à des informations supplémentaires pour détecter d'éventuels marchands de sommeil. axe, la commission a approuvé le renforcement des sanctions contre les marchands de sommeil. Au regard des coûts induits par la mise en place des procédures de permis de louer et de diviser, la commission a estimé plus logique que ce soient les collectivités qui bénéficient du produit des amendes. En contrepartie, ces mêmes collectivités ne pourront prélever de frais pour le traitement des demandes du permis de louer.

en adéquation avec les besoins. Chacun en a bien conscience, la réponse aux difficultés rencontrées ne relève pas toujours du niveau législatif. La lutte contre l'habitat indigne nécessite que les différents acteurs, collectivités territoriales comme État, se mobilisent fortement pour dépister l'habitat indigne, engager les procédures administratives appropriées et, surtout, assurer le suivi des mesures prescrites. Il s'agit d'une demande très forte des élus que nous avons rencontrés. En effet, si le préfet ne prononce pas les sanctions en matière de permis de louer, si la justice ne poursuit pas les marchands de sommeil, si les directions départementales des finances publiques ne se retournent pas contre les propriétaires défaillants pour récupérer les sommes engagées par les élus au titre des travaux d'office, les pouvoirs publics perdent toute crédibilité en la matière. Outre une mobilisation de l'ensemble des acteurs, la lutte contre l'habitat indigne suppose des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux. De ce point de vue, le dispositif APL accession est un outil essentiel de la politique de lutte contre l'habitat indigne. Chacun a pu constater les effets dévastateurs de sa suppression sur les programmes de rénovation de l'habitat indigne, tout particulièrement en outre-mer. Mais, au-delà des moyens financiers, il faut d'abord et avant tout convaincre les propriétaires de rénover leur bien, entretenir les toitures, protéger les murs extérieurs. Le parcours de rénovation énergétique performante- le PREP le PREP -est un outil intéressant à cet égard, qu'il faut bien sûr encourager. Sous le bénéfice de ces observations, je vous propose d'adopter le texte tel que la commission l'a modifié.

pour enrichir le texte initial de la proposition de loi que nous avions examinée ici même il y a quelques mois. Je veux tout d'abord saluer et remercier pour leur travail M. le sénateur Bruno Gilles, Mme le rapporteur, ainsi que l'ensemble des sénateurs de la commission

depuis deux ans avec le plan « Initiative copropriétés », la relance du programme de rénovation urbaine ou les améliorations apportées par le projet de loi ÉLAN, autant de sujets sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir.

à Marseille pour rencontrer les habitants et accompagner les sinistrés, et pour m'assurer que tous les acteurs, services et opérateurs de l'État, collectivités, se mobilisent pour gérer les suites immédiates de l'effondrement des immeubles

notamment la caserne du Muy à proximité du centre-ville. Nous allons bientôt finaliser avec la métropole et la ville de Marseille de nouveaux outils qui permettront d'accélérer la rénovation du centre-ville. Je pense à cette société de portage que nous cofinancerons- l'État entrera à son capital -ou à la mise en place d'un plan partenarial que nous développerons localement.

que vous avez adoptées dans le cadre de la loi ÉLAN. Sur le plan pénal, par exemple, la circulaire insiste sur le renforcement de la collaboration entre les services instructeurs et les parquets.

des objectifs chiffrés, discutés avec les élus locaux, par exemple sur le nombre d'arrêtés à prendre, sur le nombre de bâtiments évalués comme indignes, insalubres ou indécents.

est nécessaire d'augmenter le montant des amendes en cas de manquement à l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable à la location et de faire en sorte que ces sommes soient affectées aux collectivités locales,

Toutefois, je n'étais pas favorable à la transformation de la procédure actuelle d'accord tacite de la collectivité au bout d'un mois de silence en un refus tacite au bout de deux mois de silence

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 5 mars dernier, nous avons examiné la proposition de loi de Bruno Gilles et, considérant qu'elle pouvait être complétée, nous l'avons renvoyée en commission. Il est vrai que le drame de Marseille avait révélé l'urgence de mesures adaptées et rapidement applicables, car la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux concerne tous nos territoires,

Contextualiser la question de l'habitat insalubre renvoie à la politique du logement. Or le Gouvernement, malheureusement, persiste à ne pas écouter les alertes répétées. Alors que la reprise était engagée pour atteindre en 2017 le seuil des 500 000 logements construits, dont près d'un tiers de logements sociaux, les résultats se sont dégradés

Les raisons de ce revirement, nous les connaissons, à commencer par l'explosion du coût du foncier- il faut une politique foncière. S'y ajoutent une réduction drastique des ressources du logement social- la clause de revoyure ne nous satisfait pas -, une stratégie de vente massive du patrimoine HLM, une hausse des loyers, une précarisation accrue des publics les plus fragiles, la suppression de l'APL accession, sur nous reviendrons, le relèvement du taux de TVA à 10 % pour les opérations de construction de logements sociaux et le désengagement de l'État des aides à la pierre. Dans nos rencontres, les associations et les acteurs du logement nous ont également fait part de leurs craintes quant à la mise en application de la loi ÉLAN, par exemple, monsieur le ministre, sur l'obligation d'installer un ascenseur au-delà de deux étages.

; prévoir que le propriétaire fera deux offres de relogement, au lieu d'une ; passer l'indemnité représentative des frais de relogement d'un an à dix-huit mois de loyer.

qu'il doit y avoir un comité de suivi et de veille des ventes de logements sociaux associant les parlementaires. C'est une mesure essentielle en termes de prévention, de même que le rétablissement de l'APL accession. Clarification et simplification, notamment des polices, participent aussi de cette efficacité. Mais, alors que l'on attendait plutôt le Gouvernement sur le sujet, c'est Mme le rapporteur Dominique Estrosi Sassone qui a réalisé cet énorme travail ! La création d'une police spéciale consacrée au logement insalubre avec une autorité unique qui respecte la responsabilité des maires, comme la reprise par Mme le rapporteur de notre amendement tendant à rectifier la situation de l'occupant d'un bien présentant un danger grave et immédiat, ainsi que l'obligation faite au maire de saisir le tribunal d'instance pour qu'un syndic professionnel soit désigné sous un mois Comme le soulignait la présidente Sophie Primas, cette lutte nécessite une coordination entre pouvoirs publics sur le terrain et des moyens financiers suffisants ; à défaut, c'est leur crédibilité qui est en jeu,

L'habitat informel y est très développé, avec des taux de pauvreté oscillant entre 19 % en Guadeloupe et 44 % en Guyane ! Cette lutte passe, enfin, par le renforcement de la lutte contre les marchands de sommeil. Les collectivités territoriales doivent effectivement bénéficier des produits des amendes et les associations de lutte contre l'habitat indigne pouvoir agir en justice. Il est anormal que les maires se substituent en proposant trois offres, alors que les marchands de sommeil ne doivent en faire qu'une, fréquemment dans un lieu où personne ne veut aller ! J'ajoute, comme le rappelait Marc Daunis, qu'il est souhaitable que nous trouvions un point d'équilibre pour l'affectation des biens confisqués aux marchands de sommeil, regrettant que notre amendement visant à réaffecter ces biens au logement social ait été frappé

le drame de Marseille n'est que la partie visible d'un mal que nous ne parvenons pas à éradiquer, malgré la volonté des législateurs, des collectivités locales, des associations et de tous les acteurs participant à la lutte contre l'habitat insalubre et en péril. Il doit marquer un tournant dans notre façon de traiter le logement indigne. Cela semble être le cas, puisque le nombre d'arrêtés de péril a récemment connu une accélération et que certaines collectivités territoriales se sont pleinement engagées dans les limites de leurs moyens. L'État se doit de les accompagner. La situation de nombreux ménages, qu'il est complexe de détecter, emporte des conséquences graves et irréversibles sur l'ensemble de leurs conditions d'existence, notamment sur leur santé et, en particulier, celle des enfants. L'habitat dégradé recouvre plusieurs réalités : des propriétaires- occupants ou bailleurs -qui ne peuvent pas se permettre de rénover leur bien ou méconnaissent les aides auxquelles ils ont droit jusqu'aux marchands de sommeil qui font fortune en exploitant la vulnérabilité des occupants.

Rappelons-le, les propriétaires peuvent bénéficier des aides de l'ANAH ; en dernier recours, ils peuvent vendre le bien. Pourtant, l'arsenal répressif n'a cessé de s'étoffer. La loi ÉLAN du 23 novembre 2018 reflète la volonté du Gouvernement d'aller plus loin, en complétant les peines complémentaires obligatoires, avec la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction et l'interdiction d'acheter un bien immobilier à d'autres fins que l'occupation personnelle pour une durée maximale de dix ans. Elle atteint ainsi le patrimoine du marchand de sommeil, afin qu'il n'en use plus aux mêmes fins. Le nouveau cas d'expropriation selon la procédure simplifiée pour les logements faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter, proposé par l'auteur de la proposition de loi, va également dans ce sens. Plus d'une vingtaine de comportements sont réprimés en matière d'habitat indigne au titre du code pénal, du code de la santé publique et du code de la construction et de l'habitation. Faut-il encore renforcer la palette d'outils pour lutter contre les marchands de sommeil ?

J'espère que la circulaire du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l'habitat indigne, circulaire à destination des magistrats, marquera une évolution dans les condamnations. Ainsi, cette politique, comme bien d'autres, est victime de sa complexité. Le travail de notre rapporteur, que je tiens à féliciter, apporte une harmonisation bienvenue des procédures relatives à l'habitat insalubre et en péril, quelle que soit l'autorité compétente. a, à ce titre, exercé autant qu'elle le pouvait un droit d'amendement de plus en plus limité par les nombreuses irrecevabilités. Pour leur part, certaines collectivités ont décidé de s'approprier l'ensemble des outils qui sont à leur disposition, notamment le permis de louer et le permis de diviser. Faut-il les généraliser ? Nous le savons, des propriétaires, que je qualifierai, par euphémisme, d'« indélicats », exercent une activité souvent dissimulée. Le renforcement des sanctions pour non-respect de ces dispositifs, prévu par la proposition de loi, est donc une bonne chose. Outre le manque de moyens humains et financiers, comment détecter les situations d'habitat indigne ? Les occupants n'osent pas dénoncer, connaissant les difficultés rencontrées pour se reloger, et les visites à domicile peuvent être vécues comme des atteintes à leur intimité. Ils préfèrent, dès lors, attendre de pouvoir changer de logement plutôt que de réclamer des travaux. Nous devons donc réfléchir à l'amélioration des signalements. C'est ce que nous avons tenté de faire, Les biens dégradés doivent faire l'objet d'un suivi constant, avec données enregistrées. L'immeuble du 65 de la rue d'Aubagne à Marseille avait été signalé, semble-t-il, depuis 1953 Bien que sa finalité soit tout autre, la mise en place du carnet numérique du logement dans l'ancien en 2025 participera à cette meilleure connaissance de l'habitat indigne. Le décret du 22 mai 2019 exigeant la vérification d'une éventuelle condamnation des acquéreurs sur les ventes aux enchères n'est pas suffisant. En effet, au regard du faible nombre de condamnations, la portée de cette mesure sera de fait assez réduite. Monsieur le ministre, la crise du logement alimente directement l'habitat dégradé. Certains propriétaires occupants, une fois le bien immobilier acheté, ne peuvent plus se permettre ni de le rénover ni d'en améliorer la performance énergétique. Le reste à charge est encore élevé. La hausse des loyers et les délais d'attente pour obtenir un logement social dans les zones tendues offrent des conditions idéales aux marchands de sommeil, dont certains ont l'impression de rendre service à leurs locataires La concentration des activités dans les métropoles avec des zones où il est impossible de se loger, d'un côté, le déclin des centres-villes et des villages ruraux dévitalisés avec des logements vacants, de l'autre, traduisent l'abandon de la politique d'aménagement du territoire de ces trente dernières années.

après le drame de Marseille et plusieurs mois de travaux importants de la commission des affaires économiques, constitue un signal positif dans le traitement de l'habitat insalubre et dangereux.

Le traitement de ces plaies prend trop de temps, car notre loi est trop faible. Les causes de ces délais sont l'impécuniosité des propriétaires, les biens en déshérence, les syndics défaillants, les procédures trop longues et trop complexes, les difficultés à se substituer aux propriétaires ... La présente proposition de loi, dont l'ambition a été relevée par Mme le rapporteur, répond à toutes ces attentes. Si l'on demande aux collectivités locales d'en faire toujours plus dans ce domaine- permis de louer, permis de diviser, recrutement d'agents pour aller vérifier la salubrité des appartements, etc. -, tout cela suppose des moyens C'est pourquoi je me réjouis que la commission des affaires économiques ait accepté d'intégrer à son texte l'amendement que j'avais déjà déposé lors de la première lecture de la proposition de loi : il s'agit de rendre les travaux relatifs à l'habitat en péril éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux, Dans les plus petites communes, il arrive que des propriétaires laissent leur maison à l'abandon pour des raisons diverses- indivisions, éloignement, manque de moyens. Lorsque le maire a connaissance de désordres affectant un logement susceptible de provoquer un danger pour la sécurité des occupants ou des riverains, il notifie au propriétaire la procédure de péril. Cependant, lorsque le propriétaire est défaillant, la commune n'a que très rarement les moyens de s'y substituer dans certains cas, elle peut compter sur l'accompagnement de l'ANAH, mais celui-ci se limite aux immeubles à usage de logement. Faute de certitude en matière de recouvrement des dépenses, les maires hésitent donc parfois à engager les procédures nécessaires pour mettre fin aux situations de péril. de péril. Le recours à la DETR serait un outil supplémentaire, particulièrement utile en milieu rural. L'État ne doit pas fermer les yeux sur la détérioration de ces logements. Il doit être cohérent et allouer les moyens nécessaires. En conclusion, le groupe Union centriste votera en faveur de cette proposition de loi, telle que remaniée. Il serait bon néanmoins, monsieur le ministre, que des mesures d'ordre budgétaire puissent accompagner la prévention de l'habitat insalubre et, donc, la rénovation des logements. Sans moyens et sans prévention, nous ne ferons que « courir » après l'insalubrité, sans la combattre. Je laisse ma collègue Nadia Sollogoub compléter utilement mes propos dans quelques minutes. La parole

notre collègue rapporteur Dominique Estrosi Sassone et l'ensemble de la commission des affaires économiques, présidée par Sophie Primas, ont réalisé sur ce texte. Ce travail a permis d'étoffer et de compléter de façon pertinente la proposition de loi initiale de notre collègue Bruno Gilles. cela ne résout pas tout, mais, au moins, cela a le mérite de mettre sur la table des questions depuis trop longtemps restées sans réponse concrète. La lutte contre le logement insalubre est un sujet complexe aux facteurs multiples, un sujet nécessitant une analyse en profondeur pour trouver des solutions adaptées aux spécificités de chaque situation et de chaque territoire. Bien sûr, les enjeux du logement insalubre en zone urbaine ne sont pas les mêmes que dans les zones rurales. Dans ma région, les Hauts-de-France, pour des raisons historiques et économiques, on compte un nombre élevé de logements indignes, occupés par une population en grande précarité. Selon un récent rapport de la Fondation Abbé Pierre, 200 000 logements du parc privé y sont considérés comme potentiellement indignes. C'est beaucoup trop ! Je voudrais d'ailleurs saluer l'action de toutes les associations s'engageant au quotidien pour accompagner et aider ces foyers modestes. Ces associations réalisent un travail formidable, qu'il convient de reconnaître, accompagnant bien souvent les collectivités engagées sur le sujet. Je l'avais déjà évoqué lors de nos discussions en février dernier, le volet préventif doit être traité avec la même importance que le volet répressif. En ce sens, je me félicite du rapport qui complète utilement la proposition de loi, avec plusieurs mesures permettant de mieux anticiper les situations de logement insalubre. Concernant le diagnostic technique global, je considère toutefois que le délai proposé est trop court. je proposerai un amendement tendant à le rendre obligatoire pour les copropriétés de plus de vingt ans. Les dispositions visant à clarifier, simplifier et accélérer les procédures en matière de traitement de l'habitat insalubre ou dangereux vont également dans le bon sens. Il faut que cela soit complété et cohérent avec les mesures à venir du Gouvernement. Il faut aussi bien s'interroger sur l'autorité la plus compétente pour exercer le pouvoir de police du logement : la réponse pourra être différente selon les territoires. Le renforcement des sanctions proposé est une bonne chose. Il est pertinent qu'il soit accompagné de contrôles plus fréquents, de délais de procédure plus courts et de moyens humains et financiers appropriés. La prévention et la sanction sont deux éléments clés pour lutter contre le logement insalubre. Il faut aussi comprendre pourquoi les travaux de rénovation n'ont pas été réalisés. Les sanctions s'imposent si l'on fait face à des marchands de sommeil mal intentionnés, profitant de situations fragiles, ce que la loi ÉLAN envisageait de faire. Dans le cas de propriétaires occupants, il faut veiller à les accompagner au mieux, financièrement et administrativement, dans les travaux à réaliser. De nombreux dispositifs existent, encore faut-il qu'ils soient efficaces et connus L'Agence nationale de l'habitat joue un rôle essentiel en la matière. Dans le cadre de son programme « Habiter mieux », auquel plus de 530 000 propriétaires occupants sont éligibles, plus de 6 800 logements ont été rénovés en 2018, avec 62 millions d'euros d'aides distribuées. Le Gouvernement doit lui affecter des moyens à la hauteur des enjeux et mieux communiquer sur ces soutiens financiers. Le rôle des collectivités territoriales est primordial dans la lutte contre l'habitat indigne. Sous l'égide de grands principes ou de politiques nationales et avec l'appui d'administrations et d'agences, les agglomérations et les communes mettent en place les actions concrètes sur le terrain. C'est une prise de conscience générale que nous devons saluer à Roubaix, Saint-Omer, Amiens, Dunkerque ou Lille, je sais que les collectivités des Hauts-de-France innovent et expérimentent sur ce sujet, avec la mise en place de permis de louer, de permis de diviser ou l'intervention d'inspecteurs de salubrité, par exemple. Toutes ces initiatives doivent être soutenues et étendues dans tous nos territoires urbains et ruraux. Le renforcement du rôle des collectivités exige de leur donner les moyens nécessaires et un cadre légal leur offrant des outils pertinents pour agir.

un logement décent doit être une priorité de tous les pouvoirs publics tant il touche à la façon dont on considère notre société, ses valeurs et ses fondements.

Bien souvent, les personnes qui y vivent ont pour environnement l'humidité, l'amiante, le plomb et la promiscuité de leurs proches. La plupart d'entre eux sont victimes de marchands de sommeil. Les situations de détresse face au mal-logement sont multiples. Certains de nos enfants grandissent dans des logements si exigus qu'ils finissent par accuser un retard de développement à long terme. Face à cette rupture d'égalité, notre devoir de parlementaires est de garantir à chacun un droit à la dignité dans son logement. Le Gouvernement, grâce à votre action, monsieur le ministre, travaille ardemment à la résolution de cette question, notamment par la stratégie de lutte contre le mal-logement qu'il a engagée dès le début du quinquennat. À cet égard, je tiens à saluer trois mesures qui ont été prises et permettront d'accélérer la construction de logements là où nous en avons le plus besoin : le doublement du budget de renouvellement urbain, l'abattement fiscal pour la vente de terrains en zone tendue et, enfin, l'encadrement des recours contre les permis de construire. Cette proposition de loi, dont notre collègue Bruno Gilles est à l'origine, s'inscrit dans le même objectif global, en s'attaquant à la problématique du mal-logement : elle vise ainsi à lutter contre l'activité des marchands de sommeil. À ce stade, notre groupe soutient l'ensemble des mesures proposées. Ce texte a été patiemment amélioré après son renvoi à la commission. Nous tenons, à ce titre, à remercier la rapporteur Dominique Estrosi Sassone pour son travail d'approfondissement. Je souhaite également saluer le travail de notre collègue député Guillaume Vuilletet, qui mène une mission en ce moment sur le mal-logement. Pour lutter contre les marchands de sommeil, nous nous accordons à dire que les collectivités sont les mieux placées. Placer l'autorité de contrôle et de sanction au plus près des marchands de sommeil est la bonne stratégie. Le maire et le président d'EPCI sont ceux qui connaissent le mieux les problématiques de leurs territoires en matière de mal-logement. On ne pourra plus laisser perdurer une situation de mal-logement un an après que le bien aura été déclaré insalubre : il faudra trouver une solution dans les trois mois. Enfin, s'il faut contrôler les locations en amont, il faut aussi pouvoir sanctionner plus efficacement en aval et punir ceux qui s'enrichissent en louant un logement indigne. En aggravant les sanctions administratives encourues en cas de non-respect du permis de louer, nous sanctionnerons plus rapidement et plus efficacement. En permettant aux associations de se constituer partie civile pour poursuivre les marchands de sommeil, nous permettrons qu'ils soient plus facilement condamnés. Enfin, dans l'espoir de nourrir nos débats futurs, permettez-moi de formuler ces quelques remarques. Nous devrons veiller à ne pas oublier les propriétaires mal-logés, car c'est aussi un aspect du mal-logement. C'est par exemple le cas des logements peu onéreux, qu'il faut rénover pour les rendre habitables. Certains n'ont jamais les moyens d'assumer la totalité des rénovations nécessaires et se trouvent endettés et coincés dans ces logements insalubres. Par ailleurs, il existe des logements qui ne sont pas directement insalubres, mais qui le deviennent dès lors qu'ils sont occupés par un trop grand nombre de personnes. Ce n'est pas un phénomène mineur puisque la Fondation Abbé Pierre estime à 2,8 millions le nombre de personnes concernées. Pour conclure, je veux rappeler que la part de la dépense que les ménages consacrent au logement n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années : il est impératif de rendre les ménages capables de financer des logements à proximité des bassins d'emploi. Il faut pour cela contenir le prix de l'immobilier ; il faut construire plus Sans cela, les ménages continueront d'être pris en tenaille entre la concentration de l'emploi dans les métropoles et la hausse des prix de l'immobilier dans ces bassins d'emploi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous revoici quatre mois plus tard afin de débattre de cette proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux. Nous étions plusieurs à le souligner à l'époque, l'émotion suscitée par l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne avait conduit très justement notre collègue Bruno Gilles à déposer cette proposition de loi.

En effet, si nous voulons faire de bonnes lois, il faut prendre le temps de les travailler soigneusement. Avec la baisse du nombre de parlementaires annoncée, je crains que la situation n'aille en s'aggravant dans les années à venir. Pour en revenir au débat qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais rappeler qu'à cette heure-ci, à la suite de l'évacuation des 311 immeubles après ces tragiques événements, 223 ménages sont encore à reloger, soit un peu moins de 500 personnes, la preuve s'il en fallait que du chemin reste à faire. Du chemin que nous devons combler grâce à cette proposition de loi, car, à l'échelle nationale, plus de 400 000 logements seraient insalubres. Et je veux rappeler ici que l'insalubrité des logements n'est pas seulement l'apanage des villes : elle est aussi très présente dans nos communes rurales, déjà touchées par le fléau des « volets fermés Pour lutter, les collectivités doivent être accompagnées et nous devons leur donner les leviers afin de répondre à cet enjeu qui recoupe des enjeux nationaux de politique pénale liés à la difficulté de poursuivre les marchands de sommeil et de protéger les victimes, mais également la garantie du droit au logement, qui, je vous le rappelle une nouvelle fois, est une compétence de l'État, notamment au travers du dispositif du droit au logement opposable. Nous devons faire preuve d'ambition pour ce texte en favorisant les capacités de contrôle et d'intervention des collectivités territoriales. Nous devons aussi accélérer les réponses aux situations d'insalubrité et de dangerosité des immeubles en abaissant les délais de visite des agents attestant de l'insalubrité. Enfin, nous devons être intransigeants avec les marchands de sommeil en aggravant les sanctions administratives encourues en cas de manquement à l'obligation de déclaration de mise en location ou à celle de disposer d'un « permis de louer »- un dispositif qui n'a d'ailleurs pas tenu ses promesses et qu'il conviendrait de retravailler pour le rendre réellement et pleinement efficace. Mais une vraie politique sans vrais moyens demeurera impuissante. Je souhaite rappeler que l'ANAH, qui joue un rôle prépondérant pour la réhabilitation des logements, a longtemps vu ses financements diminuer, faisant craindre même une cessation de paiement. Son financement par le « 1 % logement » a traduit un désengagement de l'État de ses missions. Les politiques publiques des dernières années ne font qu'alimenter ces phénomènes de dégradation de l'habitat à grands coups de coupes budgétaires et de libéralisation. L'attaque frontale contre le logement social et l'assèchement de son financement, conjuguée à l'absence de régulation du parc privé, a conduit à ces dérives. Monsieur le ministre, nous n'allons pas reprendre ici les débats de la loi ÉLAN. Comme je l'avais dit il y a quelques mois, le décalage entre l'offre et la demande est tel qu'aujourd'hui les aspirants locataires se voient obligés d'accepter des logements à n'importe quel prix et dans n'importe quelle condition pour ne pas se retrouver à la rue. Parallèlement, les petits propriétaires n'ont le plus souvent pas les moyens de réhabiliter leur logement, ce qui constitue dans beaucoup d'endroits en région un potentiel de développement de l'habitat insalubre important, notamment dans les centres-bourgs. Dans ce contexte, le dispositif de revitalisation des centres-bourgs doit jouer son rôle sur cette question. Enfin, je souhaitais rappeler que trop de personnes ne sont pas au courant non plus des aides auxquelles elles peuvent avoir accès. À ce propos, comment se fait-il que les aides existantes soient aujourd'hui majoritairement destinées aux propriétaires, alors que l'on sait que la grande majorité des ménages précaires demeurent des locataires ? Comme je l'ai déjà dit, de nombreuses associations demandent aujourd'hui un véritable plan Marshall de la rénovation. Nous considérons que, pour répondre à cet enjeu, il convient, certes,

Il convient, surtout, de réorienter la politique publique du logement pour non seulement produire l'offre nécessaire de logements accessibles, mais également engager une politique de réhabilitation de grande envergure. Dans ce cadre-là, l'État doit jouer son rôle afin de permettre de trouver de nouvelles sources de financement pour répondre à cet enjeu et éviter de nouveaux drames. En l'état, nous voterons cette proposition de loi de notre collègue Bruno Gilles

Nombreux sont ceux qui, en apprenant la nouvelle dans leur journal, ont eu une pensée pour un bâtiment qui, ils le savent, montre des signes de fragilité. Nous pouvons être satisfaits de cette proposition de loi de mon collègue Bruno Gilles, car, si je redoute la qualité des textes votés sous le coup de l'émotion, le temps de la réflexion nous a été donné et je salue ici la décision de renvoi en commission qui avait été prise. Je remercie Mme la présidente de la commission Ces événements doivent nous ramener à nos responsabilités, celles de législateurs. En effet, partout en France, 450 000 logements pourraient être concernés par ce texte. À Marseille- et vous l'entendez, c'est une ville que je connais bien -, la ville, sur l'initiative de son maire, avait engagé, en 2005 déjà, plus de 200 millions d'euros,

Dans le cadre de la lutte contre l'habitat insalubre aussi, ce sont plusieurs quartiers qui avaient fait l'objet d'opérations de résorption. Et bien sûr, il y a eu les projets de rénovation urbaine et les plans successifs depuis plus de quinze ans, mais cela n'a pas suffi. Dans de nombreuses villes, l'habitat est ancien et majoritairement privé. L'intervention publique doit alors se confronter à des réglementations protectrices de la propriété privée et, au-delà des moyens financiers alloués, les procédures sont longues, trop longues, tant interviennent de nombreux acteurs. Dans le drame qui est arrivé, il y avait une procédure en cours depuis quatre ans. Aujourd'hui, nous devons adapter notre réglementation. Oui, nous devons renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des maires, élus de terrain s'il en est ! Oui, nous devons accélérer les réponses aux situations d'insalubrité et de dangerosité ! Oui, nous devons renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil Notre État croule sous cette administration toujours plus centralisée et on lui reproche légitimement cette lenteur, voire cette déconnexion, mais nous pouvons également- et heureusement -compter sur les maires qui, finalement, ne souhaitent qu'une chose : pouvoir agir. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de leur témoigner, une fois encore, notre confiance. Un maire n'est ni un agent administratif ni un bouc émissaire : il est un décideur politique légitime et pleinement compétent sur son territoire. Mes chers collègues, dans ce domaine comme dans tant d'autres, donnons aux maires de France les moyens de porter les responsabilités que l'on fait peser sur eux. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre.

que les morts de la rue d'Aubagne ne sont pas morts pour rien et que chacun prendra sa part de responsabilité. Pendant sept mois- et

Ainsi, quelques mois après la loi ÉLAN, il nous faut déjà aller encore plus loin dans la réflexion sur la qualité de notre parc immobilier national et la prévention de sa dégradation. L'objet de ce texte est d'élargir l'éventail des dispositifs en matière de prévention. Je remercie son auteur de cette initiative, ainsi que Mme la rapporteur et la commission pour avoir renforcé le texte. Lors de son premier examen, j'avais, avec mon expérience de maire d'un village de 1 500 habitants, proposé des amendements destinés à traiter de l'habitat individuel, abandonné et dangereux, que les communes de petite taille ne peuvent assumer, faute d'expertise et de budget spécifique. Il existe en effet dans nos territoires des « verrues », dégradées, abandonnées, dangereuses, qui sont pour les élus des casse-têtes insolubles. Le maire doit écrire et formaliser des mises en demeure à destination des propriétaires. Mais que faire dans le cas des successions avec plusieurs héritiers qui ne s'accordent pas, des propriétaires qui se séparent en abandonnant les lieux, chacun des protagonistes renvoyant ensuite vers l'autre ? Que faire dans le cas de propriétaires partis pour l'étranger, introuvables, insolvables ou simplement indélicats ? Les démarches et injonctions restent lettre morte. On ne sait parfois même plus à qui s'adresser. Les mois, les années passent, et le risque existe, car, même si le bien n'est pas habité- et il peut arriver qu'il le soit, les squats n'existant pas qu'en ville qui peut empêcher les enfants ou les rôdeurs d'accéder à des bâtisses abandonnées ? Et je ne parle pas du cas où le bâtiment menace la voie publique ou la propriété voisine. Alors arrive le jour où, la solution étant définitivement enlisée et le risque aggravé, il faut engager une procédure de péril imminent. Voici ce que dit la loi le maire qui a connaissance de tels faits peut, de sa propre initiative, engager une procédure de péril. Il doit saisir le tribunal administratif afin qu'il désigne un expert chargé, dans les vingt-quatre heures, de constater ou non le péril imminent. Mais qui paie l'expert ? Ces dépenses, par définition non prévues, sont rédhibitoires pour beaucoup de petites collectivités au budget très contraint. Si, grâce à l'adoption de l'amendement de ma collègue Sylvie Vermeillet, la DETR doit pouvoir venir en aide aux collectivités pour les travaux, rien n'est prévu pour les frais d'expertise.

alerte donc, monsieur le ministre, sur le frein technique et financier que constituent les indispensables expertises. Si mes propositions ne sont pas les bonnes, alors il faut en trouver d'autres. Il serait inadmissible que la lutte contre l'habitat dangereux et la prévention du risque se fasse à deux vitesses : d'une part, dans les zones d'habitat urbain tendu, où les procédures de prévention seront heureusement renforcées, et, d'autre part, en zone rurale, où les procédures de mise en sécurité resteraient définitivement inaccessibles. La parole

Dans une France qui est la cinquième puissance économique mondiale, cet état de fait nous interpelle et nous oblige à agir. Alors oui, il faut renforcer les capacités de contrôle et d'intervention des communes et des EPCI en matière de logements insalubres ou dangereux L'auteur de ce texte, Bruno Gilles, nous invite à prendre le taureau par les cornes. Mme la rapporteur, Dominique Estrosi Sassone, avec la commission des affaires économiques, a complété ce texte pour s'assurer que les réponses soient juridiquement et techniquement les plus pertinentes. Bruno Gilles nous propose, dans les zones d'habitat dégradé, de soumettre à autorisation préalable toutes les opérations tendant à diviser un logement en plusieurs, car le droit actuel ne prévoit cette possibilité qu'en cas de travaux. Or le propre des marchands de sommeil, c'est précisément de ne pas réaliser de travaux Aussi, il faut détacher l'autorisation préalable de la réalisation de travaux et l'exiger en toutes circonstances. Ce texte modifie également les conditions de délivrance par le maire ou le président d'EPCI du « permis de louer » un logement lorsque la commune l'a instauré. le silence gardé pendant un mois par le maire sur une demande de « permis de louer » vaut délivrance de cette autorisation. Il n'y a donc pas d'obligation formelle pour l'autorité saisie de s'assurer que le logement appelé à être loué ne présente pas de danger. Il faut inverser le dispositif en remplaçant la décision implicite d'acceptation par une décision implicite de refus. Le texte vise aussi à permettre au maire ou au président d'EPCI de consulter le casier judiciaire d'une personne qui sollicite un « permis de louer » ou un permis de diviser un logement dans les zones à risques au regard de l'insalubrité. Il propose encore de simplifier, dans le respect du droit de propriété, l'expropriation en raison de l'insalubrité ou de la dangerosité des immeubles. Actuellement, la loi n'envisage l'insalubrité ou la dangerosité comme une cause

Ainsi, le texte réduit la durée maximale d'habitation, abaisse de trois mois à un mois le délai imparti pour qu'un agent se rende sur place lorsqu'un citoyen saisit l'administration. Il renforce l'efficacité des sanctions contre les marchands de sommeil et aggrave les sanctions administratives. Bruno Gilles a tiré les conséquences de la forte réticence des occupants des logements loués par des marchands de sommeil. Il complète ainsi la faculté ouverte aux associations de se constituer Mme la rapporteur, Dominique Estrosi Sassone, dont on connaît l'expertise en matière de logement et le souci d'efficacité et d'efficience, a apporté beaucoup d'améliorations au texte un diagnostic technique obligatoire pour les copropriétés de plus de quinze ans ; la possibilité pour les syndics de faire des signalements ; la création d'une police spéciale du logement en cas d'insalubrité sur le modèle de celle existant en cas de péril, même si, selon les cas, cette police ne relève pas de la même autorité- maire pour le péril, préfet pour l'insalubrité, mais même procédure la présence obligatoire d'un syndic professionnel pour la durée de l'arrêté de péril ou d'insalubrité. Elle s'est efforcée de renforcer le rôle des collectivités dans cette lutte grâce à plusieurs dispositions : la mise en place d'un droit de priorité au profit des collectivités territoriales pour bénéficier du bien exproprié ; la création d'un nouveau cas d'expropriation ; le versement du produit des amendes prononcées aux collectivités qui assumeront le traitement des demandes du « permis de louer » ; la dispense pour le bailleur de demander un « permis de louer » lorsqu'il aura déjà obtenu une autorisation expresse depuis moins d'un an. Enfin, et surtout, elle a prévu des sanctions plus lourdes contre les marchands de sommeil. Il ne s'agit pas d'un texte pour se donner bonne conscience après le drame de Marseille.

Bouc émissaire, ce dernier subit souvent la frustration de l'impuissance, puis l'injustice de la mise en cause. Alors, donnons au maire les prérogatives lui permettant d'agir, pour ne plus avoir à subir. La discussion générale est close.

de la commission, avons été reçus, partout sur le territoire, par des élus qui mettent beaucoup de moyens et d'énergie pour lutter contre

quand il existe entre 450 000 et 600 000 logements insalubres en France, dont 70 000 dans les outre-mer, la lutte contre l'habitat insalubre est un impératif national. national. C'est pourquoi nous soutenons les mesures de la proposition de loi, telles que l'accélération des procédures et le renforcement du contrôle et des sanctions. Je reprends volontiers ses propos pour évoquer la situation du département de l'Aude.

à n'importe quel prix, en zones de marché tendu, voire division abusive de logements ou de maisons dans un objectif de rentabilisation maximale. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ajouterai que près de 20 000 logements sont potentiellement indignes dans l'Aude, plus de 41 000 personnes étant concernées. Ce parc de logements indignes est en constante augmentation ; deux ménages sur cinq sont des propriétaires occupants et les ménages de plus de 60 ans sont particulièrement concernés, avec 37 % des logements potentiellement indignes près de 5 % des résidences principales dans l'Aude sont dans les catégories cadastrales les plus médiocres, contre 3,8 % dans toute l'Occitanie : pas de WC, absence fréquente de locaux d'hygiène, qualité de construction vétuste. Cela représente près de 8 300 logements, qui constituent le noyau dur que doivent cibler les actions de lutte contre l'habitat indigne. Enfin, 40 % de ces logements

Les propositions de notre collègue Bruno Gilles et le travail de grande qualité fait par la commission, tout particulièrement par Mme Estrosi Sassone, méritent d'être soutenus. Pour autant, je ne voudrais pas que nous nous fassions d'illusions excessives, car, vu l'ampleur des problèmes, je crains qu'il ne suffise pas d'améliorer techniquement les dispositifs législatifs existant. de la discussion du projet de loi de finances, des besoins financiers. Mme Estrosi Sassone a justement mis en exergue un certain nombre de décisions qui auraient pu être prises si les procédures parlementaires ne bridaient pas nos initiatives, comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, j'y insiste, rien n'est possible sans la volonté politique des élus et sans la persévérante détermination de l'État. Il se trouve que, en 2002, j'ai signé, au nom du Gouvernement, un protocole d'éradication de l'habitat insalubre

est-il que l'État, puisque c'est de sa compétence, n'a pas eu la persévérance de mettre en oeuvre le protocole, et la ville de Marseille a manifestement considéré que le problème n'était pas aussi essentiel que cela pour interpeller l'État.

puisqu'il permet d'informer les copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en oeuvre dans le cadre d'un plan pluriannuel. pluriannuel. Il est préférable de prévoir un diagnostic technique global obligatoire pour les immeubles construits depuis plus de vingt ans et soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Vous avez ouvert aux organismes vendeurs la possibilité de mettre en place un dispositif de mise en copropriété différée. C'est une bonne chose pour sécuriser les accédants. Toutefois, nous pensons qu'il faut aller plus loin. La vente des logements sociaux ne doit pas mettre en danger la situation financière des ménages ou la qualité du bâti vendu ni produire de nouvelles copropriétés dégradées, alors que

Ainsi, le plan de vente prévu par la CUS pourrait comporter, pour chaque immeuble destiné à la vente, un état descriptif de l'état du bâti et des équipements mentionnant les gros travaux réalisés les cinq dernières années et les travaux d'amélioration que l'organisme prévoit d'engager le cas échéant. Cette mesure de transparence nous paraît essentielle pour éclairer toutes les parties prenantes de la vente de logements sociaux et prévenir la dégradation de copropriétés nouvelles. Je profite de cet amendement, monsieur le ministre, pour vous demander de mettre en place un comité de suivi et de veille des ventes de logements sociaux et d'y associer les élus locaux et les parlementaires. Permettez-moi de revenir sur un point précédent. Pour l'avoir vécu, je peux témoigner que l'opération de Bron Terraillon,

soit directement intégré à la convention d'utilité sociale que chaque office HLM doit conclure pour faire part de sa stratégie patrimoniale. On le sait bien et cela a été rappelé, pour combattre l'habitat indigne, plus on agit en amont,

descriptif du bâti et des équipements ainsi que les travaux réalisés au cours des cinq dernières années et les travaux d'amélioration que le bailleur social prévoit d'engager.

des travaux et des charges de copropriété, non pas des cinq dernières années comme vous le proposez, mais des deux dernières années, doit être communiqué. Enfin, comme vous le proposez, la liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun à entreprendre ainsi qu'une évaluation du montant global des travaux et des quotes-parts qui seraient imputables

D'après le code de la sécurité sociale, le logement doit réunir les caractéristiques de décence pour ouvrir droit aux aides au logement. Dans les faits, ces critères ne sont vérifiés que si les occupants font l'objet d'un contrôle, ce qui reste très peu probable. Ainsi, pour faire respecter le droit, les caisses d'allocations familiales, les CAF, ne peuvent se reposer que sur l'attestation de loyer, seule pièce justificative requise concernant le logement. Elles ont mis en place une grille d'auto-évaluation pour inciter les locataires à déclarer un logement potentiellement indécent. Or ces derniers n'ont pas intérêt à dénoncer leurs conditions de logement s'ils veulent obtenir les aides. Le seul moyen qui permettrait aux CAF de détecter un logement non décent serait d'être destinataires du contrat de location, qui contient un dossier de diagnostic technique et un état des lieux.

Nombreux sont les marchands de sommeil qui s'assurent un niveau élevé de rentabilité de leur logement grâce aux aides financières de la caisse d'allocations familiales. Depuis 2014, la loi ALUR donne le droit à la caisse d'allocations familiales de suspendre jusqu'à dix-huit mois toutes aides financières au logement si un logement est considéré comme insalubre ou indécent afin d'obliger les propriétaires à réaliser les travaux nécessaires. Malheureusement, les moyens alloués à la CAF pour contrôler ces logements ne sont pas assez importants. Par conséquent, les cas de procédures de suspension allant à leur terme se font rares. Il s'agit d'un problème majeur pour les victimes des marchands de sommeil. Lorsque leur plainte à la CAF n'aboutit pas à une suspension des aides, les occupants font malheureusement souvent l'objet de pressions et de menaces de la part de leur propriétaire. Il est donc important qu'un état des lieux soit réalisé et que le recours à cette disposition soit plus largement étendu.

que l'insalubrité d'un logement ne soit pas une situation isolée et qu'elle concerne en réalité l'ensemble de l'immeuble. Cet amendement a un objet pragmatique : il s'agit de permettre à l'agent missionné par le maire ou le représentant de l'État, à la suite du signalement d'un particulier, de constater dans un document séparé les désordres qu'il a pu observer lors de son déplacement sur le bâti en général. Cela permettra aux autorités compétentes de mieux apprécier la situation et d'envisager des mesures, y compris en l'absence de signalement exprès des occupants.

L'article 193 de la loi ÉLAN a introduit l'obligation pour l'agent immobilier et pour le syndic de copropriété de saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une atteinte à la dignité humaine ou un non-respect d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. De son côté, le notaire a uniquement l'obligation de signaler la non-conclusion de la vente d'un bien immobilier lorsque la personne a déjà été condamnée. Les marchands de sommeil se fournissent dans le vivier de biens à rénover, notamment lors des ventes aux enchères, raison pour laquelle la loi ÉLAN a également posé l'interdiction pour une personne ayant fait l'objet d'une condamnation d'acquérir un bien par ce biais. Or l'efficacité de ces deux derniers dispositifs repose sur la condamnation, encore rare, du propriétaire. Afin de repérer les biens potentiellement insalubres ou en péril, le présent amendement vise à prévoir que le notaire chargé d'établir l'acte authentique signale ces faits aux autorités compétentes. Ces dernières pourront apporter une réponse plus rapide en prescrivant des mesures ou des travaux.

: La parole est à M. Éric Gold. La loi ÉLAN a rendu obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction, ou de l'indemnité d'expropriation, ainsi que l'interdiction d'acquérir des nouveaux biens pendant une durée maximale de dix ans. Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé de la peine d'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que celle-ci a été utilisée pour commettre l'infraction en matière d'habitat insalubre ou dangereux. Il s'agit ainsi d'empêcher le propriétaire concerné de continuer à alimenter facilement,

plus tolérante avec le propriétaire non occupant qui, de mauvaise foi, ne rénove pas son patrimoine immobilier. Cet amendement d'appel vise donc à prévoir que le juge ne puisse pas écarter l'application des peines complémentaires lorsque le bien insalubre ou en péril n'est pas occupé par le propriétaire. Quel est l'avis de la commission ?

aux copropriétés dégradées sont assez peu opérationnels. Cet amendement vise à renforcer leur pouvoir en amont afin de leur permettre d'avoir une vision d'ensemble des copropriétés placées sous administration provisoire par le biais d'outils dont les modalités de fonctionnement et d'accès resteront à définir.

Gold. Pour résoudre un problème d'habitat insalubre, il faut dans un premier temps poser un diagnostic, puis solliciter des aides financières souvent illisibles et complexes, et enfin engager et superviser les artisans chargés de réaliser les travaux, tout en gérant un relogement parfois inévitable.

Le recours à une personne référente, mise à disposition par la collectivité, permettrait de sortir de l'insalubrité et de l'insécurité un certain nombre de locataires. Il s'agit par ailleurs à la fois d'une question de santé publique et d'écologie. En aidant les propriétaires, nous favorisons les travaux d'isolation des bâtiments, lesquels permettent ensuite de réduire la consommation d'énergie. Quel

Il pourrait également être intéressant d'intervenir là aussi en amont, sans attendre que le bâti soit dans un état pouvant être dangereux pour ses occupants, notamment en simplifiant la procédure de mise en oeuvre d'un état de carence. telle simplification se doit bien entendu de respecter les principes du droit de propriété, mais la temporalité est un enjeu important dans ce type de situation. Cet amendement vise donc à imposer un délai plus court pour la remise du rapport d'expertise lorsque la procédure est enclenchée. Par ailleurs, il faut souligner que l'expert désigné pour constater la situation de la copropriété rencontre en pratique des difficultés pour obtenir les comptes auprès des syndics.

l'intention des auteurs de cet amendement. Sur le plan formel, la disposition est insérée dans un article sur le permis de louer, alors qu'elle aborde un tout autre sujet. Sur le fond, je m'interroge sur la mise en oeuvre opérationnelle du dispositif, l'amendement ne précisant pas les copropriétés dégradées concernées- s'agira-t-il des copropriétés sous administration provisoire, des copropriétés soumises à un plan de sauvegarde ?- de sauvegarde ?- ni les pouvoirs de ce comité. Actuellement, les élus sont systématiquement informés des différentes mesures prises concernant les copropriétés dégradées. En cas de difficultés et d'impayés importants, le maire est informé de la saisine du tribunal. Si le juge désigne un mandataire, le maire reçoit le rapport du mandataire. Il en va de même en cas de nomination d'un administrateur Si la copropriété nécessite la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde, le préfet met en place une commission pour effectuer un bilan de la situation et faire des propositions.

à défaut de rendre obligatoire le permis de louer, dans les zones délimitées au regard de l'objectif de lutte contre l'habitat indigne. Conscients que les marchands de sommeil ne procèdent pas en principe à la déclaration de location ou à une demande de permis de louer, nous espérons que le renforcement des peines prévues dans la proposition de loi les incitera davantage à le faire. Cette généralisation reste moins contraignante que celle du permis de louer et permettrait aux collectivités locales compétentes en matière d'habitat d'être informées des biens immobiliers potentiellement indignes mis en location. En outre, le propriétaire devant remettre un récépissé de la déclaration de mise en location pour bénéficier du tiers payant des aides personnalisées au logement, cette mesure constitue également un outil d'information pour les caisses d'allocations familiales. Quel est l'avis de la commission ? La ? La commission émet un avis défavorable. Il paraît souhaitable de garder de la souplesse en la matière et de laisser les collectivités décider si elles souhaitent ou non mettre en place la déclaration de mise en location.

Mme Annie Guillemot. Depuis la loi ALUR, l'EPCI ou la commune peuvent mettre en place ce que l'on appelle communément le « permis de louer » sur des périmètres d'habitation présentant une proportion importante d'habitat dégradé et dans l'objectif de lutter contre l'habitat indigne. Cette autorisation préalable doit être sollicitée avant chaque mise en location. En revanche, le dispositif actuel n'oblige pas le propriétaire à renouveler l'autorisation préalable en cas de reconduction du bail. S'agissant de zones et d'immeubles identifiés à risque, il est proposé que l'autorisation préalable ne soit pas un blanc-seing donné au propriétaire pendant toute la durée d'occupation d'un ménage dont le bail peut se renouveler par tacite reconduction. Notre amendement instaure une durée de validité du permis de louer.

tous les trois ans. Le dispositif proposé ne règle pas la situation du locataire si le permis de louer n'est pas attribué à l'issue des trois ans.

contraire au principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile. Enfin, le permis de louer a été conçu comme un outil à utiliser en amont de la mise en location. Lorsque le locataire est déjà dans les lieux, les polices spéciales du péril, de l'insalubrité et la saisine du juge en cas de non-décence doivent automatiquement prendre le relais. J'ajoute que la CAF peut conserver les APL pour obliger le bailleur à réaliser les travaux pour rendre le logement décent.

monsieur le ministre,

est à Mme Annie Guillemot. Les associations que nous avons rencontrées comme Droit au logement ou la Fondation Abbé Pierre, qui suivent les familles, nous ont fait part de dossiers particulièrement difficiles avec des enfants atteints de troubles psychologiques

Je souhaite à ce stade revenir sur la très grande avancée que nous avons adoptée en commission, et que le groupe socialiste avait défendue, consistant à permettre au maire d'utiliser ses pouvoirs de police générale et de prendre toute disposition pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d'instruction du dossier. La prise d'un arrêté de péril ou d'insalubrité prend bien souvent trop de temps, laissant les familles dans des situations d'extrême précarité. Cette possibilité ouverte au maire pourra également s'avérer utile dans la phase d'instruction, les propriétaires indélicats exerçant une pression accrue contre leurs victimes pour faire respecter une loi du silence assortie de menaces, de violences, de chantages, ou encore de voies de fait. fait. Nous proposons de consacrer un chapitre à la protection des occupants d'habitat indigne qui subissent ces pressions. En effet, les marchands de sommeil ne doutent de rien et certains n'ont pas hésité à solliciter du juge des référés la résiliation du bail pour défaut de paiement au cours d'une

et éventuellement de leur recours en indemnisation. Pour renforcer la protection des occupants, même si nous en connaissons la difficulté, il est proposé d'intégrer au sein du code de la construction et de l'habitation une présomption de bonne foi de l'occupant. Le droit au relogement des occupants d'habitat indigne serait ainsi mis en oeuvre, sauf en cas de mauvaise foi avérée

sur le propriétaire en matière de relogement lorsqu'est prononcée une interdiction d'habiter les lieux en application d'un arrêté d'insalubrité ou de péril. Le propriétaire doit ainsi reloger le locataire, le sous-locataire et l'occupant de bonne foi. S'il ne peut les reloger, il doit verser un an de loyer aux pouvoirs publics, qui doivent assurer le relogement. Vous proposez dans votre amendement d'inverser le principe et d'étendre la charge pesant sur les propriétaires avec une réserve, celle de la mauvaise foi avérée. Nos collègues évoquent également les cas où le bail a été résilié et où se pose la question de savoir si l'on doit reloger ou non l'occupant. Si, lors d'une demande en justice pour résilier le bail, les locataires démontrent au juge l'existence de l'arrêté de péril ou d'insalubrité justifiant la cessation de paiement des loyers, le bail ne peut pas être résilié

Mme Samia Ghali. Cet amendement vise à enrichir le principe de « logement adapté aux besoins et aux possibilités » déjà inscrit dans la loi, afin qu'il réponde à l'ensemble des problématiques que rencontrent les personnes délogées pendant leur relogement.

De ce fait, inscrire dans la loi et encadrer les critères de relogement des personnes victimes de l'habitat insalubre est essentiel. Les personnes déplacées ne sont pas responsables de l'avis de péril

qui n'a pas choisi d'habiter dans un logement voire un immeuble en péril et qui doit en subir les conséquences pendant de longs mois, voire quelques années.

indélicat qui doit s'occuper du relogement des occupants. Nous pensons qu'il faut frapper plus fort. Il y a un paradoxe à confier le relogement du locataire victime à son propriétaire délictueux, notamment en cas de relogement définitif, au risque de laisser les occupants dans la spirale de l'habitat indigne. S'agissant d'un logement définitif, et pour limiter le risque de retour vers un autre logement insalubre, notre amendement prévoit que le propriétaire fera deux offres de relogement, au lieu d'une actuellement, répondant aux besoins et aux ressources du locataire ou de l'occupant.

qui n'interviennent qu'après avoir constaté la défaillance du propriétaire. Le contentieux sur le fait de savoir si l'offre du propriétaire est adaptée ou non risque de doubler, retardant

de vote. Sur cette question de l'APL accession, le Président de la République a dit des choses extrêmement précises pendant le grand débat.

est en train d'être expérimentée. On a demandé au ministère des outre-mer de nous aider à faire cette expérimentation à une échelle un plus importante. Celle-ci va commencer en Guyane,

avec ses absences, ses vacances parlementaires, etc. En septembre, nous serons obnubilés par la réforme constitutionnelle.

Monsieur le ministre,

avec une aide au foncier de la métropole de Lyon et de la ville de Bron, d'acquérir. Aujourd'hui, elles ne le peuvent plus. L'APL accession, qui ne coûte que 50 millions d'euros, permettait à des familles, dont le logement était démoli dans le cadre des programmes de

L'indemnité représentative des frais engagés pour le relogement en cas de défaillance du propriétaire est limitée actuellement à un an de loyer prévisionnel. Il est proposé de renforcer l'indemnisation due par les propriétaires indélicats ou marchands de sommeil. souhaitons en effet porter l'indemnité de relogement à dix-huit mois de loyer au lieu d'un an, et ce sans aucun état d'âme. Cet amendement vise également à permettre aux maires d'imposer au propriétaire ou à l'exploitant défaillant de s'acquitter d'un droit de réservation auprès d'un organisme d'HLM. Finalement, c'est comme une réquisition. Il n'y a pas de raison

vous demandez d'abord que, en l'absence de critères, le choix relève du maire ou du préfet. Je pense que cela peut être sujet à contentieux. Je m'interroge ensuite sur le fait d'imposer un droit de réservation,

Quel est l'avis du Gouvernement ?